les questions de défense seront abordées au travers de deux axes : d'une part, le renforcement des capacités de production de notre industrie de défense européenne, d'autre part, la préparation du sommet de l'Organisation

le Conseil européen devrait revenir sur la question des migrations après le terrible naufrage au large de la Grèce et les récentes avancées enregistrées sur le pacte sur la migration Comme vous le savez, sur l'ensemble de ces sujets, la situation évolue tous les jours, et les positions que je vous exposerai ce soir sont encore susceptibles d'être ajustées, notamment dans le cadre des concertations conduites entre Européens.

mois la possibilité de la paix- une paix choisie, donc durable. Un nouveau seuil a été franchi avec la destruction partielle du barrage de Kakhovka. Il s'agit bien entendu d'un acte grave, d'un acte inexcusable et odieux, qui aura des conséquences durables sur la vie de milliers d'Ukrainiens déjà meurtris par la guerre et qui ont dû être évacués. De plus, cet acte met en danger l'environnement et l'avenir des récoltes. Il menace aussi de façon irresponsable la sécurité de la centrale nucléaire civile de Zaporijia. Évidemment, la Russie cherche à semer le doute sur l'origine de ce sabotage, mais nous ne devons pas perdre de vue un fait simple : c'est elle, et elle seule, qui porte la responsabilité de cette situation. C'est elle qui a engagé cette guerre, c'est elle qui bombarde, c'est elle qui tue, c'est elle qui détruit les infrastructures civiles, au service d'un projet aussi impérialiste qu'illégal. Face à cette situation, les chefs d'État et de gouvernement rappelleront donc leur engagement à soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, y compris en assurant un soutien financier de long terme.

les chefs d'État et de gouvernement reviendront sur les actions engagées par l'Union européenne (UE) et par les États membres en matière de lutte contre l'impunité des crimes internationaux commis en Ukraine et en matière de recours aux actifs russes gelés et immobilisés. Enfin, le Conseil européen réaffirmera la perspective européenne de l'Ukraine et de la Moldavie. Il saluera les progrès réalisés vers l'adhésion à l'UE sur sur la base de l'évaluation orale que rendra la Commission cette semaine, à l'occasion du conseil Affaires générales informel de Stockholm auquel je participerai demain et après-demain. Le Président de la République a été très clair à l'occasion de son discours à Bratislava : la question pour nous n'est pas de savoir si nous devons élargir l'UE- nous y avons répondu il y a un an -ni quand nous devons le faire- pour nous, le plus vite possible -, mais bien comment. Permettez-moi

Nicolae Popescu a d'ailleurs eu l'occasion de répéter la semaine dernière au bureau de la commission des affaires européennes combien le soutien de la France était apprécié à Chisinau. Deuxièmement, une large partie du Conseil européen sera consacrée aux questions économiques, dans leurs dimensions

à l'. Les chefs d'État et de gouvernement débattront surtout de la stratégie de sécurité économique européenne. Lors de son discours à La Haye, à l'institut Nexus, le Président de la République a esquissé les contours de cette nouvelle doctrine, dont l'objectif est d'assurer pleinement notre souveraineté. Elle repose sur cinq piliers complémentaires. Le premier pilier Nous devons continuer d'innover, de réformer et de renforcer nos systèmes éducatifs et de formation. Nous devons aussi approfondir le marché unique pour favoriser l'émergence d'acteurs économiques européens plus forts. Le deuxième pilier concerne la politique industrielle. Je serai contente d'entendre que la France a joué un rôle clé pour faire progresser la politique industrielle européenne : ce concept n'est désormais plus un tabou. L'Europe doit continuer en ce sens pour asseoir son leadership industriel.

Il s'agit de protéger nos entreprises contre les actions hostiles et les distorsions de concurrence, de réduire les dépendances stratégiques de l'UE, de protéger notre propriété intellectuelle et de mobiliser nos instruments de défense commerciale.

pour que les producteurs européens soient soumis aux mêmes règles de production que les entreprises qui produisent à l'extérieur de l'Union

Le Conseil européen donnera des orientations pour sa mise en oeuvre, qui devra s'appuyer sur des analyses concrètes de nos dépendances et de nos besoins. Nous veillerons également au respect des compétences nationales pour les aspects les plus sensibles. sensibles. Troisièmement, ces enjeux de sécurité économique ont un lien direct avec l'Europe de la défense, qui sera également à l'agenda du Conseil européen. effet, si nous voulons continuer à soutenir l'Ukraine dans la durée, il faut passer dès maintenant à une économie de guerre européenne. Il faut donc renforcer les capacités de production de l'industrie de défense de l'Union européenne et mettre en oeuvre rapidement les propositions de la Commission dans ce domaine.

Sénat. Le Conseil européen devra aussi permettre de dessiner les grandes lignes de l'avenir de la coopération entre l'Union européenne et l'Otan, dans l'esprit de la troisième déclaration conjointe sur la coopération du 10 janvier 2023. Comme vous le savez, cette déclaration souligne l'apport pour la sécurité transatlantique d'une défense européenne renforcée.

nous sommes complètement déterminés à poursuivre, avec responsabilité et solidarité, le travail engagé avec nos partenaires européens sur les questions migratoires. Cette tragédie doit nous rappeler l'importance de la coopération entre Européens et avec les pays tiers en matière de sauvetage en mer et de lutte contre les réseaux de passeurs. la réforme de notre système européen d'asile et de migration, nous venons de franchir une étape très importante : le Conseil a trouvé un accord sur les principaux textes du pacte sur la migration et l'asile : ils contiennent chacun une mesure phare de notre futur cadre européen commun en matière de solidarité et de responsabilité. Je pense que c'est un résultat dont nous pouvons collectivement être fiers. Nous sommes bien plus proches désormais d'une réponse européenne sur cette question, alors que les réponses exclusivement nationales se sont évidemment soldées par des échecs. Néanmoins, ces succès internes ne doivent pas nous faire oublier le nécessaire travail que nous devons mener sur les aspects externes. Il faut à présent intensifier le renforcement de nos partenariats avec les pays tiers et avec les pays d'origine, afin de traiter les causes profondes des migrations et de prévenir les départs.

la Chine, le Conseil européen sera l'occasion d'une discussion stratégique, qui s'inscrira dans la continuité de la discussion entre ministres des affaires étrangères tenue lors du Gymnich du 12 mai me semble que l'on peut en retenir une certaine convergence de vues entre États membres, au moins sur la pertinence du triptyque européen : « partenaire, concurrent commercial et rival systémique peut aussi en retenir le besoin d'actualiser notre stratégie, afin de tenir compte de la montée en puissance de la dimension de rivalité systémique.

et renforcer les instruments européens de lutte contre les pratiques commerciales déloyales et abusives, comme je l'évoquais tout à l'heure dans le cadre de notre doctrine de sécurité économique. En parallèle, nous devons bien sûr maintenir le dialogue avec Pékin sur les enjeux globaux. La participation du Premier ministre chinois, Li Qiang, au sommet de Paris pour un nouveau pacte financier mondial, ces jours-ci, en est d'ailleurs l'illustration.

nous souhaitons rappeler que les questions des droits de l'Homme, de la démocratie et de l'État de droit restent fondamentales. Ces thématiques sont centrales dans la relation avec de nombreux pays latino-américains, et il conviendra d'aborder ouvertement ces sujets. La situation à Haïti sera également mise en avant par la France et d'autres partenaires, européens comme latino-américains : nous devons agir collectivement et rapidement pour le rétablissement de la sécurité et d'un cadre démocratique. ailleurs, les perspectives de coopération ouvertes par le devraient constituer des livrables importants du sommet avec un agenda d'investissement dans la région qui est en cours d'élaboration. Je pense que nous ne pourrons pas réduire notre partenariat économique aux accords commerciaux. Cet agenda d'investissements sera donc extrêmement important. La victoire de Recep Tayyip Erdogan et de son parti aux dernières élections présidentielle et législatives a ouvert une nouvelle phase en Turquie. Je tiens d'ailleurs à saluer le sénateur Leconte pour sa participation à la mission d'observation électorale dans ce pays, au titre de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe Maintenant que le scrutin est derrière nous, il sera utile que nous ayons une discussion plus approfondie à vingt-sept. La Turquie est évidemment un acteur important de notre voisinage : il est par conséquent essentiel de poursuivre le dialogue et de maintenir la coopération avec elle sur les sujets d'intérêt partagé dans le contexte international et régional dégradé que nous connaissons. Au-delà de ces élections, il faut aussi rappeler que tout réengagement de l'Union européenne à l'égard d'Ankara doit être subordonné à la capacité des autorités turques à remplir les conditions fixées par le Conseil européen en mars et en juin 2021, ainsi qu'à prendre des mesures concrètes sur les questions de politique étrangère les plus urgentes, s'agissant notamment de l'adhésion rapide de la Suède à l'Otan l'Otan et du contournement des sanctions adoptées en réaction à l'agression russe contre l'Ukraine. Il est essentiel que nous restions unis et que nous soyons parfaitement clairs quant à nos attentes à l'égard de la Turquie. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà, en quelques mots, les enjeux de ce Conseil européen. Je ne doute pas que vos questions me fourniront l'occasion de revenir plus en détail sur l'un ou l'autre de ces points. La parole

Cette LPM doit être inscrite dans le cadre global de la réaction déterminée et unie des pays européens face au retour de la guerre sur notre continent. Dans un contexte inédit de « réveil géopolitique de l'Europe la programmation des dépenses militaires de la France est un aspect essentiel de notre crédibilité comme acteur stratégique sur le continent. Le projet de LPM que nous avons examiné tend à rappeler que la France constitue « un acteur clé » de la défense de l'Europe et qu'elle doit y assumer des « responsabilités particulières de vue capacitaire, la constitution d'une base industrielle et technologique de défense (BITD) européenne réactive, robuste et souveraine est un objectif que nous portons de longue date. Il faut espérer que les menaces grandissantes qui pèsent sur notre sécurité commune provoquent une prise de conscience collective et rapide. Seule une volonté politique partagée et clairement affirmée nous permettra de mener à bien nos grands projets capacitaires à développer à l'échelle européenne. Je pense en particulier au projet de système de combat aérien du futur (Scaf), que nous élaborons actuellement avec l'Allemagne et l'Espagne. Ces travaux de développement menés en commun pour élaborer les technologies militaires qui équiperont nos armées demain sont essentiels. De plus, madame la secrétaire d'État, nous devons nous organiser dès à présent pour répondre dans l'urgence au défi humanitaire, diplomatique, opérationnel, mais aussi logistique, que représente notre soutien collectif à l'effort de guerre ukrainien. L'Union européenne et ses membres ont démontré depuis le 24 février 2022 leur capacité à soutenir l'Ukraine dans la durée et et sans que l'unité européenne soit remise en cause, ce qui est extrêmement important. Cette unité fait notre force, et j'insiste sur l'importance de ne pas céder à la tentation d'une division artificielle, dont nos compétiteurs et nos adversaires seraient évidemment les premiers bénéficiaires.

Si nous souhaitons aider l'Ukraine, nous ne désirons pas, en revanche, que la Commission européenne centralise les informations des entreprises de la BITD pour les utiliser à sa guise. Nous faisons face ici à des sujets qui qui touchent au coeur de la souveraineté nationale. Par ailleurs, le commissaire Thierry Breton a insisté sur sa volonté d'une adoption rapide de ce programme de financement d'urgence. Alors que le Parlement européen a voté en faveur de ce plan le 1 juin dernier, nous vous demandons, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement défende clairement nos positions sur ce point. Notre commission soutient le renforcement de la défense européenne, mais selon des modalités pragmatiques qui n'empiètent pas sur notre souveraineté dans ce dans ce domaine éminemment sensible. En matière de défense, efficacité opérationnelle est synonyme de subsidiarité. Enfin, j'évoquerai brièvement un sujet qui concerne notre politique de commerce extérieur. En août 2019, le Président de la République a fait état de son opposition à la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et Mercosur au regard du risque de concurrence déloyale qu'il pourrait faire peser sur certains de nos producteurs. À la fin de l'année 2021, le Président a réaffirmé son opposition au traité dans son état actuel au motif qu'il est incompatible avec notre agenda climatique et de biodiversité. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a adopté une résolution invitant le Gouvernement à réitérer son opposition à l'adoption du traité et à son application partielle. Pourtant, le voyage récent de la présidente Ursula von der Leyen en Amérique du Sud aussi bien que les perspectives dessinées pour la présidence espagnole du Conseil de l'Union européenne au semestre prochain ont renforcé l'attention portée à ce traité et à l'hypothèse de sa ratification par l'Union européenne. Dans ce contexte, madame la secrétaire d'État, ma question est la suivante quelle position la France défendra-t-elle au Conseil européen sur ce dossier ? Quelles sont vos priorités pour mettre en oeuvre une politique commerciale européenne qui assure la défense de nos producteurs en cohérence avec nos objectifs climatiques ? La parole est à M. le

D'une part, la hausse des taux d'intérêt, qui découle de l'inflation, remet en cause les hypothèses de remboursement des intérêts du plan de relance et risque, par conséquent, d'affecter des programmes budgétaires déjà approuvés. D'autre part, la guerre en Ukraine a fait émerger de nouvelles dépenses en matière de sécurité alimentaire et énergétique, de prise en charge des réfugiés ou encore de défense. De plus, une révision ambitieuse du CFP impliquerait de nouveaux besoins de financement. En ce sens, la Commission a annoncé qu'elle joindrait à cette réforme un second panier de nouvelles ressources propres. Parmi ces dernières, la Commission européenne pourrait notamment présenter un nouveau cadre pour la fiscalité des entreprises. En tout état de cause, les retards pris dans la mise en oeuvre des nouvelles ressources propres du premier panier, en particulier le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, m'incitent à rester prudent face à ces annonces. Dans ce contexte, madame la secrétaire d'État, pourriez-vous nous préciser la position du Gouvernement sur une éventuelle révision du cadre financier pluriannuel ? sujet de son financement, l'adoption de nouvelles ressources propres à moyen terme vous paraît-elle réaliste ? En ce qui concerne mon second sujet, la réunion du Conseil européen devrait être l'occasion d'un échange de vues sur la réforme de la gouvernance économique européenne. Elle intervient alors que la Commission européenne a présenté, le 26 avril dernier, ses initiatives de réforme de la gouvernance budgétaire. Les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance connaissent des critiques qui sont anciennes. Elles n'ont pas permis de prévenir des trajectoires fortement divergentes en matière d'endettement public entre les États membres. De plus, elles ont pu constituer un frein à la mise en oeuvre de politiques publiques de soutien à la croissance économique et n'ont pas contribué à accentuer l'investissement public. Les propositions formulées par la Commission européenne viennent achever un débat ouvert par la suspension du pacte de stabilité et de croissance opérée lors de la crise sanitaire. Sans revenir sur la règle de limitation des déficits et de l'endettement à respectivement 3 % et 60 % du PIB, la Commission européenne propose notamment de maintenir le cadre commun de surveillance en rendant plus automatique la mise en oeuvre des sanctions. que les États s'engagent sur des trajectoires pluriannuelles de moyen terme en décrivant leurs cibles budgétaires et les réformes et investissements envisagés. de tenir compte des investissements prévus pour la transition écologique, pour le numérique et pour la défense. Enfin, elle invite à différencier les objectifs prévus pour chacun des États en fonction de la situation de leurs finances publiques. Certaines de ces propositions me semblent aller dans le sens d'une amélioration souhaitable du cadre existant. En premier lieu, l'individualisation des trajectoires des États devrait permettre une meilleure appropriation nationale des règles budgétaires. En second lieu, je ne puis qu'approuver la prise en compte des investissements dans le suivi des trajectoires nationales. Si la Commission européenne n'a pas retenu une différenciation de la dette selon sa nature, sa proposition vise à préserver l'investissement des efforts de de redressement des comptes publics à venir et à accroître les dépenses favorables à la transition écologique. Ces dépenses d'avenir sont indispensables, alors que la réalisation de nos objectifs de transition impliquera un effort d'investissement

Par ailleurs, de quelle manière le Gouvernement souhaite-t-il se saisir de ce cadre favorable à l'investissement pour accélérer nos efforts en matière de transition écologique ? La parole

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous débattons ce soir très en amont de la prochaine réunion du Conseil européen, alors même que son ordre du jour n'est pas encore publié sur la page internet qui est lui Cela nourrit nos interrogations sur la méthode suivie dans les travaux de notre assemblée en matière européenne. Grâce à la secrétaire générale du Conseil, que la commission des affaires européennes a auditionnée récemment, nous avons toutefois pu obtenir quelques indications le prochain Conseil européen devrait principalement parler d'Ukraine, de défense, d'économie, de relations extérieures et d'enjeux migratoires. À n'en pas douter, la priorité du Conseil européen sera de faire le point sur la contre-offensive ukrainienne. Ce qui est en jeu, c'est la sécurité du continent. À ce titre, le soutien de l'Union européenne ne saurait faillir. La solidarité non plus, et l'on peut à cet égard s'inquiéter de la divergence franco-allemande qui se creuse ostensiblement en matière de défense, notamment en ce qui concerne le bouclier antiaérien. Le Conseil européen, en mars dernier, a pointé du doigt l'urgence d'un approvisionnement suffisant de l'Ukraine en munitions à ce stade du conflit. C'est pourquoi la Commission européenne, le mois dernier, a proposé un texte destiné à accélérer la production de munitions dans l'Union, mais aussi à assurer leur disponibilité, en surveillant les stocks et leur localisation. Autant nous soutenons l'urgence d'une relocalisation de la production de munitions sur le sol européen- nous l'avons déjà appelée de nos voeux en amont du Conseil européen de mars -, autant nous sommes inquiets du caractère très intrusif des pouvoirs que la Commission européenne entend se donner à cet effet, dans un domaine éminemment régalien, sur lequel l'information est très sensible et échappe d'ailleurs largement aux parlementaires que nous sommes. Madame la secrétaire permanents (Coreper) qui devrait examiner ce texte déjà adopté en urgence au Parlement européen, nous tenons à appeler les autorités françaises à la plus grande vigilance sur ce dossier stratégique. J'ai proposé au président de la commission des affaires étrangères, Christian Cambon, de formaliser ensemble cet appel par un courrier officiel à la Première ministre, auquel je souhaite associer les rapporteurs de la commission des affaires européennes qui nous ont alertés sur le sujet, nos collègues Gisèle Jourda et Dominique de Legge. Concernant l'Ukraine, le Conseil européen de la fin juin sera informé du rapport que la Commission publiera demain et qui évaluera les progrès des réformes attendues en matière de justice et de lutte contre la corruption et le blanchiment, en Ukraine comme en Moldavie. À cet égard, l'interdiction du parti de l'oligarque prorusse Ilan Shor, décidée hier par le Conseil constitutionnel de Moldavie, constitue une avancée indéniable. la route est longue vers l'élargissement, même si l'Ukraine réclame d'ouvrir sans délai les négociations pour son adhésion et que la Géorgie entend bien, avant la fin de l'année, se voir reconnaître à son tour le statut de pays candidat. Nous ne devons pas oublier que, parmi les critères à considérer avant tout élargissement, l'un concerne l'Union européenne elle-même. Il s'agit de sa capacité d'absorption dans quelle mesure l'Union européenne est-elle capable de se maintenir comme union de paix si elle intègre des États qui sont en guerre, qui abritent des conflits gelés, comme en Transnistrie, ou qui n'ont pas résolu leurs contentieux de voisinage-

Même si je doute qu'il aille aussi loin, le Conseil européen ne pourra pas, lors de sa prochaine réunion, ignorer les questions immédiates que soulève déjà la révision à mi-parcours des perspectives financières de l'Union,

dont l'impact n'est pas sérieusement évalué, ils se trouvent menacés de subir la concurrence déloyale du Mercosur, avec lequel la Commission européenne et la prochaine présidence espagnole du Conseil semblent pressées de conclure un accord. Doivent-ils aussi craindre que le budget de la politique agricole commune ne fasse les frais des priorités que la Commission européenne a fait valoir aujourd'hui même, à savoir le soutien à l'Ukraine, la riposte aux subventions États-Unis et la Chine consacrent à leur économie pour en assurer la compétitivité, ou encore l'appui financier aux pays de départ pour réguler les flux migratoires ? De fait, la pression migratoire redouble en Méditerranée centrale et trop de bateaux surchargés font naufrage sous nos yeux. Les avancées enregistrées au Conseil sur le pacte sur la migration et l'asile permettent d'espérer en finir avec l'impuissance. Madame la secrétaire d'État, que peut-on attendre du prochain Conseil européen à ce sujet qui figure expressément à son ordre du jour ? Moins d'un an nous sépare des élections européennes : il n'est plus temps de tergiverser pour donner à l'Union européenne les moyens de ne pas subir l'avenir. La parole

le compte à rebours est lancé : dans moins d'un an, nous serons appelés aux urnes pour les élections du Parlement européen. Bien des bilans seront dressés dans les douze prochains mois. Les institutions européennes voudront mener à bien nombre de propositions engagées qui reflètent les promesses, mais aussi les évolutions dues aux récentes crises. Le mandat 2019-2024 est un tournant pour notre Union européenne et pour nous tous. à l'heure des premiers bilans, je crois plutôt que nous devrions continuer inlassablement d'avancer. Nous entrons dans une période de débat où la question principale est de savoir quelle Union européenne nous voulons inventer pour demain. Le 9 mai dernier, le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré qu'il souhaitait une union ouverte et renforcée. Sur certains sujets, nous sommes plutôt alignés, par exemple sur l'extension du vote à la majorité qualifiée à plusieurs domaines- encore faut-il savoir lesquels ... La fiscalité est une est une piste, mais ce n'est pas la seule. Les affaires étrangères en sont une autre. Le groupe Les Indépendants est attaché au débat sur ce sujet. L'unanimité est un frein parfois trop important pour que l'Union européenne avance correctement dans l'intérêt des citoyens européens. D'autres points développés par le chancelier font partie des nombreux désaccords des derniers mois. Il n'y a rien d'insurmontable, certes, mais nos visions divergent sur certains dossiers. Cela enrichit le débat, mais apporte aussi de nombreuses frustrations et parfois des incompréhensions. Quelques-uns des sujets que je vais aborder en sont des exemples types. Avant cela, j'aimerais formuler une remarque de forme sur le débat préalable que nous avons ce soir. Au-delà de l'heure tardive, un sujet que j'ai déjà évoqué il y a quelques mois, j'y ajouterai : « Mieux vaut tard que jamais ». Nous avons en effet reçu l'ordre du jour du Conseil européen il y a seulement quelques heures ... Le rôle des élus nationaux, particulièrement des parlementaires, dans le système européen est important. Cela ne concerne pas uniquement la subsidiarité. Nous sommes au fait de ce qui se passe sur nos territoires, de ce que vivent les Européens. Notre parole est l'amplification de la leur. Les orientations et questions dont nous nous faisons ce soir le relais sont les leurs- ne l'oublions pas ! Pour revenir sur les sujets européens, celui de l'énergie fait bien sûr partie des priorités. Pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, nous rassurer quant aux réserves en gaz pour l'hiver prochain ? La France pourra-t-elle atteindre au 1 novembre prochain ses objectifs en matière de stockage ? Le tout premier appel d'offres pour des achats groupés de gaz a été lancé début mai. Quels sont les premiers retours et quand est prévu le prochain ? Le marché intérieur de l'électricité est l'un des dossiers les plus urgents de cette fin d'année. Qu'attendez-vous du prochain Conseil européen concernant la proposition d'évolution du système et l'objectif de son adoption avant la fin de l'année ? Depuis mars dernier et les dernières conclusions du Conseil européen, notre position n'a pas changé concernant la guerre d'agression contre l'Ukraine. Je souhaite la réitérer : les responsables des crimes de guerre devront être jugés et les crimes documentés ; je pense notamment aux déportations d'enfants ukrainiens, car ce sujet reste central. Alors que l'Ukraine a lancé sa contre-offensive, pouvez-vous déjà nous indiquer où en est le prochain paquet de sanctions à l'encontre de la Russie et quelles sont ses grandes lignes ? Est-ce que le paquet est prêt à être présenté lors du Conseil dans dix jours ? Dans les dernières conclusions du Conseil européen, il a également été question des migrations. Mercredi dernier, la Méditerranée a encore été le théâtre d'un drame humain : des dizaines de personnes sont mortes noyées en espérant rejoindre le sol européen. Ces victimes viennent malheureusement allonger une liste déjà bien trop longue de plusieurs dizaines de milliers de personnes mortes dans les mêmes conditions depuis une décennie. La mer Méditerranée ne peut être un cimetière à ciel ouvert. Ce drame survient seulement quelques jours après qu'il y a eu accord en Conseil de l'Union européenne des ministres de l'intérieur sur deux principaux axes du pacte européen sur la migration et l'asile. Ce pacte est complexe à faire aboutir, et nous savons que l'objectif est une adoption avant juin prochain. Le principal mécanisme est celui qui est dit de solidarité. Comment la France envisage-t-elle sa mise en pratique entre les deux options proposées : la relocalisation des réfugiés et la compensation financière ? Comment le sujet sera-t-il abordé lors du Conseil européen ? Enfin, parce que c'est un sujet qui me préoccupe particulièrement et qu'il y a urgence, je souhaite ce soir aborder une nouvelle fois la question du cyberharcèlement. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle est un risque supplémentaire, notamment dans la création de contenus. L'Union européenne l'a bien compris, je salue le travail mené par le commissaire Thierry Breton concernant un pacte sur l'intelligence artificielle. Il est important de trouver un cadre efficace. Je sais le processus européen long et complexe, 2025 semble bien loin. Je vous encourage, madame la secrétaire d'État, ainsi que vos collègues, à faire en sorte qu'une solution efficace soit rapidement trouvée en Conseil de l'Union européenne, mais aussi au Parlement européen.

Je souhaite que nous soyons intraitables collectivement sur la bonne mise en place de ces normes, ainsi que sur leur efficacité, quitte à être très réactifs si nous observons des dysfonctionnements et des besoins de révision des règles. Nous serons nombreux au Sénat à y être très attentifs. La parole

Nous saluons donc la volonté du Gouvernement de persister à soutenir l'Ukraine par tous les moyens qui sont nécessaires. Nous continuons à porter le projet d'une défense européenne, pour que l'Europe soit autonome stratégiquement et militairement. Pour le reste, qu'en est-il aujourd'hui de notre projet européen, de notre cohésion sur les grands objectifs et de nos valeurs communes ? Ils sont- c'est leur lot -ballottés, malmenés, voire carrément reniés. Ce Conseil européen serait utile s'il contribuait à redonner vigueur à ces impératifs qui fondent notre unité. Dans nombre d'États européens, les surenchères sécuritaires prospèrent, les entraves au Pacte vert se dressent, le lobbying en faveur de la finance et du libre marché gagne du terrain, droite, voire les coalitions avec elle, se multiplient. À un an des élections européennes, nous attendons des responsables européens la clarté et la détermination nécessaires pour donner envie d'Europe en plus et en mieux. Au large de Kalamata, à proximité du Péloponnèse, c'est dès l'après-midi que Frontex a pu prendre la mesure du drame qui se nouait, qui se nouait, mais c'est à 23 heures cette nuit-là que l'embarcation abandonnée à son sort a sombré avec près de 750 personnes Ce bilan est l'un des plus lourds des dernières années ; ces dizaines et peut-être centaines de morts viennent s'ajouter aux 1 300 autres recensés depuis le début de 2023. Bien sûr, la culpabilité première revient aux trafiquants d'êtres humains, profiteurs de celles et ceux qui fuient la misère, la guerre et, de plus en plus, un dérèglement climatique invivable. Bien sûr, cette culpabilité est première, elle ne décharge pas pour autant les politiques européennes de leur lourde part de responsabilité. Il faut, hélas, le dire clairement : ces morts sont un peu à mettre au bilan de Frontex. En se reniant depuis tant d'années face aux discours anti-migrants, en intensifiant les politiques migratoires très restrictives, le contrôle de ses frontières, en sous-traitant à des pays où les droits humains sont bafoués, l'Europe a fait de la Méditerranée la voie migratoire la plus meurtrière au monde. monde. Si ce Conseil européen entend vraiment lutter contre cette mortalité effroyable au seuil de l'Europe, son urgence doit être d'organiser la coopération pour les sauvetages- vous venez d'en dire un mot, madame la secrétaire d'État. Or l'accord du 15 juin entre les États membres sur le pacte sur la migration et l'asile n'ouvre aucune perspective de création d'une force européenne de secours en mer. Ce nouveau drame y oblige ; c'est un impératif minimum.

Paris a totalement bloqué les choses jusqu'à ce que ses demandes sur le nucléaire soient satisfaites dans ce texte clé du Pacte vert qu'est la proposition de directive relative aux énergies renouvelables. Il a donc fallu que la Commission européenne finisse par acter « la reconnaissance du nucléaire dans l'atteinte de nos objectifs de décarbonation ». on dénonçait les manoeuvres de blocage de nos voisins allemands sur les voitures thermiques. Aujourd'hui, on les imite ! Ce lobbying déstabilise les investissements dans la décarbonation et en encourage d'autres : ainsi, hier, en Conseil des ministres européens de l'énergie, la France a soutenu la prorogation des subventions aux centrales à charbon existantes jusqu'en 2028- encore un recul ! Ce retard sur nos objectifs de décarbonation coûtera cher, tout comme le démantèlement annoncé de Fret SNCF, pour lequel le gouvernement français semble capituler avant même d'avoir mené la bataille, alors que notre cause avait des raisons solides, partagées en Europe. Plutôt que de tenir, vous consentez à en finir avec Fret SNCF. Comment la mise à la découpe de cette entreprise pourrait-elle ne pas briser le rebond ferroviaire nécessaire et ramener des camions sur les routes ? À quoi en Europe veut-on donner la priorité ? Au climat ou à la libre concurrence ? Cette question vaut également pour l'accord UE-Mercosur, tel qu'il a été conclu en 2019, que l'Assemblée nationale vient de rejeter dans une résolution. Cet accord serait une usine à dérégler le climat, à accroître la déforestation, à contaminer l'environnement, à détruire l'agriculture paysanne coloniser les terres des peuples autochtones. Le respect de l'accord de Paris et celui de nos normes sanitaires et environnementales pour tout produit agroalimentaire importé, voilà la ligne à tenir, sans pour autant couper les ponts avec l'Amérique latine. L'Union européenne peut aider à protéger l'Amazonie, en respectant ses engagements en matière de financement de l'action climatique et par ses aides en faveur des forêts des pays du Mercosur. Cela passe aussi par une directive ambitieuse Les eurodéputés ont voté un texte prometteur prévoyant un mécanisme de responsabilité civile et un accès renforcé des victimes à la justice européenne, qui a nettement élargi le champ des entreprises concernées et qui inclut le secteur financier et la chaîne de valeur aval des entreprises.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, douze ans : depuis douze ans, je prends la parole à l'occasion de chaque débat préalable au Conseil européen, ainsi qu'à l'occasion de tous les autres débats qui ont trait à l'Europe dans cet hémicycle. Ne vous méprenez pas : pour moi, c'est tout sauf un pensum ou une sinécure ! Et si je m'attelle ce soir à cet exercice pour la dernière fois, parce que j'ai fait le choix de vous quitter bientôt, c'est plus que jamais avec plaisir et passion, sans amertume aucune. Je suis Je suis né Européen sans le savoir, et c'est grâce au voir et au savoir que je le suis devenu. J'ai beaucoup parcouru l'Europe avant de devenir sénateur ; j'ai continué de le faire en l'étant, je le ferai davantage encore en ne l'étant plus. Ce continent, qui porte le beau nom d'une princesse d'Asie enlevée par Zeus, est si beau et si complexe, si riche et si fragile aussi, qu'il mérite que nous consacrions ce qui nous reste de futur personnel à tenter de préserver le sien. Mais, s'ils ont souvent la même fragilité, un être humain et un continent ne s'inscrivent évidemment pas dans la même temporalité. Dans la part de temporalité commune qui peut exister entre une personne et son territoire, c'est-à-dire entre notre histoire personnelle et l'Histoire tout court, chacun peut mesurer sa chance au regard des événements heureux qui lui ont été donnés de vivre, mais aussi au regard d'événements terribles auxquels il a eu le bonheur d'échapper. Nous sommes tous ici, dans cet hémicycle, issus de plusieurs générations qui ont eu la chance de ne pas connaître la barbarie nazie, ses cortèges de morts, de déportés et d'exactions sans nom. Cette longue paix, nous la devons bien évidemment à l'Europe, à sa patiente construction dans un cadre démocratique, en dépit des crises et soubresauts qui l'ont traversée et qui continuent de le faire. Lorsque nous en disposons depuis longtemps, la paix comme la liberté passent pour acquises au point de faire figure de non-événement. C'est une erreur, pis, une cécité, de ne pas voir que, chaque matin, lorsqu'elles se réveillent, tant de personnes dans tant d'autres parties du monde s'interrogent sur ce que la journée aura peut-être de fatal pour elles ou pour leurs proches. l'heure du retour de la guerre dans l'est de notre continent, c'est une chose que nous omettons de raconter et d'expliquer à nos enfants, car, parfois, nous n'en avons nous-mêmes plus guère conscience. l'événement européen de portée véritablement historique vécu par les générations ici représentées restera certainement la chute du mur de Berlin, la fin du rideau de fer et l'effondrement de l'URSS. Ce fut la promesse d'une aube nouvelle pour l'Europe, mais si soudaine, si bouleversante et si enthousiasmante pour les peuples du continent que nous avons omis à l'époque de mesurer pleinement les défis que cette Europe élargie poserait à plus long terme. Parce que le régime soviétique, tel un cyclope éborgné, s'était écroulé de lui-même, nous avons voulu croire à la fin de toute velléité impériale de la part de la Russie. Triste aveuglement qui n'est pas étranger à l'horrible tragédie qui secoue aujourd'hui l'Ukraine. Quand j'ai choisi il y a douze ans de devenir sénateur, plutôt que de tenter de devenir eurodéputé, j'avais la conviction profonde que c'était au plus proche de nos concitoyens qu'il fallait parler d'Europe, afin afin de la rendre audible autant que sa complexité le permet. En effet, il ne suffit pas d'être un Européen convaincu ; il convient surtout d'être un Européen convaincant, capable d'expliquer les enjeux réels qui se posent à nous dans un monde de plus en plus délicat à appréhender. Au cours de ces douze dernières années, notre Europe a connu bien des crises, au point de se demander si leur succession, désormais incessante, n'est pas devenue, bien plus que le présumé moteur franco-allemand, le coeur du réacteur de son processus d'approfondissement et sans doute, demain, de son processus d'élargissement. Ébranlée, bousculée, parfois au point de pouvoir être renversée, l'Union européenne, malgré sa plasticité de boxeur plus apte à encaisser les coups qu'à en donner, a cependant bien plus évolué durant la décennie écoulée ce cheminement vers davantage d'intégration politique ne s'est fait, pour l'essentiel, qu'en réaction aux nombreuses crises que nous avons traversées. Il serait illusoire de croire qu'il puisse en être autrement : les États membres n'acceptent de se départir d'une part de leur souveraineté nationale que, lorsqu'en lorsqu'en ultime instance, ils finissent par admettre leur incapacité à affronter seuls un défi qui les dépasse. Que cela nous plaise ou non, il ne saurait en être autrement, et le « Grand Soir constituant », rêvé par nombre d'européistes convaincus, n'a plus l'heur de convaincre et de faire espérer. Il en est ainsi, et il faut cesser de voir dans le réel l'ennemi de la politique. Le réel n'est que la matière à partir de laquelle se construisent patiemment les édifices. À la liste des sujets traités lors des Conseils européens depuis plus d'une décennie illustre bien l'évolution, certes lente, mais profonde, qui a affecté l'Union européenne au cours de la période et qui préfigure peut-être son devenir. Au début des années 2010, presque tout ce qui était débattu en Conseil renvoyait à la crise financière de 2008, à ses conséquences directes et indirectes, à la crise de l'euro et à la déflagration violente suscitée dans les pays du sud de l'Europe. Les réponses proposées renvoyaient encore et toujours au renforcement du marché unique, véritable Graal des chevaliers de la Table ronde du Conseil ... On était prêt à sacrifier la Grèce sur l'autel d'une orthodoxie qui n'avait rien de religieux, mais tout de financier. La politique extérieure de l'Union européenne, hors la multiplication effrénée d'accords de libre-échange, se limitait à quelques timides politiques de voisinage, dont, au passage, il serait bon un jour de tirer un bilan honnête et sans fard.

ans auparavant, j'étais à Zagreb, à quelques kilomètres du front, sous les pluies de tirs perdus qui tombaient sur la capitale. Au risque de passer pour un fou en France, je militais déjà activement en faveur d'un avenir européen pour ce pays. À la fin de ce séjour, notre délégation sénatoriale fut reçue par le Président de la République, Ivo Josipovic. Surprise : nous avions sympathisé vingt ans auparavant en pleine guerre, il était alors universitaire et musicologue, et nous nous étions ensuite perdus de vue au fil des ans. Le 1 juillet 2013, la Croatie devint le vingt-huitième membre de l'Union européenne. Nous ignorions à l'époque que ce serait, à ce jour, le dernier pays à rejoindre l'Europe. Nous ignorions aussi que, quelques années plus tard, un État membre de l'Union européenne prendrait la décision impensable de la quitter. L'avenir de l'Europe est souvent imprévisible, et nous sommes, particulièrement aujourd'hui, payés pour le savoir. Mais ce que je veux retenir ici, c'est que, au prix d'immenses efforts, la Croatie vient en ce début d'année de rejoindre la zone euro et l'espace Schengen. Schengen. C'est un signe d'espoir : il peut y avoir une vie européenne après la guerre. Cependant, dans la situation actuelle, avec la guerre qui fait rage en Ukraine, la question majeure que devront se poser les chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront dans quelques jours à Bruxelles est grave, extrêmement grave. ni plus ni moins que de savoir s'il peut subsister une Europe après la guerre horrible conduite par la Russie, si l'Ukraine venait à perdre celle-ci. La réponse est vraisemblablement non ! Et le poids de notre responsabilité en la matière sera immense si nous renonçons à aller plus avant dans notre soutien à Kyiv. Pour conclure sur une touche différente, je tiens à saluer très chaleureusement les trois présidents de la commission des affaires européennes qui se sont succédé depuis 2011, Simon Sutour, Jean Bizet et naturellement Jean-François Rapin, avec lesquels j'ai eu, durant ces douze années, le grand bonheur de travailler. je vous remercie

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous devons débattre ce soir de l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil européen. Cependant, le contexte économique, social et sociétal que vivent les Européens nous oblige à évoquer également d'autres questions essentielles pour lesquelles la vigilance de chacun doit être de rigueur. Depuis le début de 2021, l'inflation a vivement augmenté dans les principales économies de la zone euro. Les prix des produits alimentaires ont progressé de 15 % par rapport à 2020 et expliquent à eux seuls près de la moitié de l'inflation, pénalisant les ménages les plus modestes, qui consacrent une part importante de leur budget à l'alimentation. Une inflation élevée réduit le pouvoir d'achat des citoyens et rend de nombreuses entreprises moins compétitives ; surtout, elle a un impact disproportionné sur les personnes à faible revenu. Dans un tel contexte, les conséquences de la hausse de 0,25 point de son taux d'intérêt par la Banque centrale européenne, annoncée le 4 mai dernier, doivent être questionnées. d'abord, parce que cette hausse prive les plus modestes de l'accès au crédit et vient s'ajouter à la réduction du pouvoir d'achat des Européennes et des Européens. Ensuite, parce que, aujourd'hui, l'inflation est tirée par les superprofits, la cupidité, l'avidité. Elle est liée au maintien des marges des entreprises. La Banque centrale européenne a également émis des craintes contre cette spirale des prix « qui pourrait appauvrir tout le monde ». La question d'un contrôle temporaire des prix se pose donc pour prévenir les spirales inflationnistes de ces prix abusifs. parce que la hausse des taux d'intérêt va dégrader directement la rentabilité des opérations de rénovation énergétique des logements et des bâtiments ; elle va plus globalement détériorer la rentabilité des investissements de la transition écologique que nous devons financer. S'il faut saluer l'assouplissement des règles budgétaires proposé par la Commission européenne, l'angle mort de cette réforme demeure la question des recettes pour financer les transitions. Qui va payer pour augmenter les dépenses vitales en vue d'atténuer les émissions de CO2, réduire par là même notre dépendance aux énergies fossiles, largement importées,

Nous avons besoin d'un plan pérenne et de réponses concrètes de la Commission européenne sur ce point. Nous avons besoin d'une capacité budgétaire européenne. Nous avons besoin de justice fiscale, de taxation sur le capital et d'un prélèvement pour le marché unique, parce que, si l'on aime l'Europe, on la finance ! Le 8 juin dernier, un projet d'initiative citoyenne européenne appelant à créer un impôt européen sur les grandes fortunes a été déposé auprès de la Commission européenne par l'eurodéputée Aurore Lalucq et le président du parti socialiste de Belgique Paul Magnette. soutenus notamment par Thomas Piketty et l'ancien commissaire européen hongrois Laszlo Andor, ainsi que par plusieurs ONG, comme Oxfam, et par des millionnaires eux-mêmes. Tous plaident pour la création d'un impôt européen sur les grandes fortunes. Partout dans le monde, les plus riches parmi les plus riches sont beaucoup moins taxés que les autres en proportion de leurs revenus, parce qu'ils bénéficient d'une fiscalité avantageuse sur le capital ou qu'ils ont la capacité de défiscaliser L'Institut des politiques publiques a montré, dans sa note en date du 6 juin dernier, que, à partir d'un certain seuil de richesse, le taux d'imposition régresse, car les profits que les ultra-riches que les ultra-riches tirent de leurs sociétés échappent au calcul de l'impôt sur le revenu. Il est temps de rétablir une fiscalité plus juste et équitable. L'économiste américain Joseph Stiglitz, lauréat du prix Nobel, avait même proposé de mettre en place un taux d'imposition mondial spécial de 70 % sur les revenus sur les revenus les plus élevés, ainsi qu'un impôt sur la fortune de 2 % à 3 %. Avec mes collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, je ne puis que relayer avec force ces propositions alors que nous plaidons, depuis plusieurs mois maintenant,

l'Union européenne. Aujourd'hui, de nombreuses organisations telles que l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae), le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), ou encore l'Agence française de développement (AFD) concluent que nous pourrons nourrir les 10 milliards d'habitants que comptera le monde en 2050. En revanche, pour ce faire, quelques conditions doivent impérativement être respectées : mettre un terme à l'accaparement des terres et les partager ; assurer le renouvellement des générations en garantissant un revenu digne à tous les paysans, partout dans le monde ; enfin, établir un commerce équitable non seulement entre les espaces ruraux et les métropoles, mais aussi entre les pays et entre les continents. Or, madame la secrétaire d'État, cet accord est archaïque tant sur le fond que sur la forme. On ne peut pas promouvoir une agriculture durable en faisant de la lutte contre le changement climatique une priorité et, dans le même temps, faire venir sa viande de l'autre bout de la planète en favorisant un modèle agricole intensif, responsable à 80 % de la destruction de la forêt amazonienne. Il s'agit non pas de militer uniquement à des fins protectionnistes, mais d'agir au nom d'une souveraineté solidaire, afin que la France affirme ses valeurs universelles tout en défendant ses propres intérêts, lesquels rejoignent en toute logique ceux de l'humanité. cet accord est un désastre pour les éleveurs et agriculteurs des deux côtés de l'Atlantique. Les importations de boeuf en provenance du Mercosur pourraient augmenter de 50 %. Ce sont 99 000 tonnes équivalent carcasse de boeuf sud-américain, potentiellement élevé aux antibiotiques, que nous importerions sans imposer de droits de douane, alors même que nous avons, à raison, banni les antibiotiques de croissance en Europe à compter du 1 janvier 2006. 2006. Comment assurer notre souveraineté alimentaire face à un accord qui menace le bien-vivre de celles et ceux qui nous nourrissent ? C'est en remettant en cause ce traité que nous pourrons, dans les conditions que j'ai exposées, nourrir les 10 milliards d'habitants attendus d'ici

Nous le considérons comme une aberration sociale et écologique. De même, le projet de réforme du marché européen de l'électricité, désormais mis dans la boucle du trilogue Commission européenne-Conseil européen-Parlement européen, nous paraît sans rapport avec les ambitions affichées initialement.

mais la mise en oeuvre de cet accord s'annonce encore très longue. En revanche, c'est aussi le moment choisi par le président Macron pour faire d'Elon Musk la nouvelle grande vedette

Les conceptions qui sont mises en avant nous semblent davantage motivées, en vérité, par une logique de guerre économique. La façon dont les relations entre l'Union mises à l'ordre du jour de ce Conseil européen en témoigne à nos yeux. Il y a quatre ans seulement, le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne publiaient une communication conjointe sur leur vision stratégique

dit-on, de relocaliser la production de technologies vertes suffisamment matures, essentielles à la décarbonation, pour lesquelles l'Europe est aujourd'hui bien trop dépendante. si la Chine produit aujourd'hui 75 % des panneaux photovoltaïques et des batteries, presque 60 % des éoliennes et 40 % des électrolyseurs

rapidement : « Dans la course qu'elle a engagée pour construire avant les autres un nouveau modèle de croissance verte, c'est-à-dire pour définir les standards de demain et établir une position forte dans les industries du futur, l'Europe prend le risque d'additionner les handicaps. Elle cumule en effet retards industriels, coût de l'énergie élevé, exposition aux fuites de carbone et volonté de ne pas s'écarter de la discipline budgétaire. Si certaines contraintes, sur les prix de l'énergie notamment, lui sont imposées par le contexte international, certaines disciplines, en particulier en matière budgétaire, résultent de ses propres décisions. » Allons-nous tirer des leçons de ces constats pour être moins belliqueux, mais plus offensifs en matière de reconquête industrielle, en poussant les feux d'un fonds souverain européen et d'un renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou en utilisant la création monétaire

maintenant l'Ukraine dans l'Otan, si nous donnions ce feu vert, alors, nous le savons tous, la frontière orientale de l'Union européenne se verrait transformée en ligne de front de l'Otan, de l'Arctique à la Méditerranée. Je ne crois pas que ce soit ainsi que nous mettrons fin à la guerre

que ce serait la voie, non pas d'une victoire rapide, mais d'une guerre longue, terriblement destructrice, coûteuse et dangereuse. La solution de rechange à la guerre devrait plutôt être la mobilisation de toutes les forces de l'Union européenne et de toutes les coalitions mondiales possibles pour des solutions politiques de paix et de sécurité. Le surarmement, la militarisation et « l'otanisation » de l'Europe ne préparent pas ce chemin-là. J'espère, madame la secrétaire d'État, qu'à Vilnius la raison demeurera assez forte pour que la France ne donne pas son feu vert à cette adhésion, qui ne réglera pas les problèmes, mais risquerait de les aggraver encore. La La parole est à M. Jean-Michel Arnaud.

La sécurité du continent renvoie évidemment à la guerre russo-ukrainienne. Oui, nous y sommes : la contre-offensive ukrainienne a débuté, comme l'a confirmé le Président de la République. L'escalade des tensions et la situation précaire à l'Est viennent mettre à l'épreuve la stabilité et la sécurité de la région européenne dans son ensemble. Le soutien apporté à l'Ukraine dans sa lutte pour la préservation de son intégrité territoriale doit se poursuivre. Le combat que mène ce pays force le respect. Le groupe Union Centriste, comme d'autres, se tient évidemment derrière le peuple ukrainien et apporte son plein soutien à nos amis qui se battent pour les valeurs de l'Union européenne. aussi à célébrer les trente ans du marché unique, qui appelle à une meilleure compétitivité de nos entreprises européennes. Si notre union économique et monétaire permet à l'Europe de demeurer une puissance commerciale mondiale, ses bénéfices n'ont pas été uniformes pour tous les États membres.

À la suite des crises successives que nous avons traversées, l'objectif d'une souveraineté économique européenne semble faire consensus. Médicaments, batteries électriques, avions propres : nombre de pistes se dessinent. Il faut s'en saisir, mais les Européens doivent aussi faire preuve de cohérence.

C'est d'autant plus dommageable que nos deux pays coopèrent sur le programme Scaf, le système de combat aérien du futur. La compétitivité européenne ne dépend donc pas uniquement de la qualité des investissements réalisés ou de l'étendue de nos innovations ; elle repose également sur leur bonne adéquation avec notre politique commerciale. Il y va de la prospérité de nos filières d'avenir, à l'instar de l'agriculture en France. Alors que les moyens financiers de la politique agricole commune ont été revus à la hausse, le Pacte vert européen prévoit une baisse de la production agricole.

dans le domaine de la transition énergétique que les États membres s'opposent actuellement. En ce qui concerne la réforme du marché de l'électricité, un point de désaccord majeur subsiste. Les Vingt-Sept se déchirent sur les modalités des contrats pour la différence, à prix garanti par l'État. Dans ce mécanisme, le producteur d'électricité doit reverser les revenus engrangés si les cours du marché de gros sont supérieurs au prix garanti, mais perçoit une compensation dans le cas contraire. La Commission européenne proposait que tout soutien public à de nouveaux investissements dans la production d'électricité décarbonée se fasse impérativement ce type de contrat. Si la France s'en réjouit, d'autres États, tels que l'Allemagne ou le Luxembourg, y sont hostiles. Madame la secrétaire d'État, que pouvez-vous nous dire sur l'état d'avancée de ces discussions importantes pour nos territoires ? Je pense à certaines TPE ou

Tel est par exemple l'objet de la plateforme de marketing digital Utiq, récemment lancée par des opérateurs français, allemand et espagnol, afin de concurrencer les géants américains. Le DSA vise

Oui, l'espace numérique est un espace public comme un autre, mais il s'agit d'un espace où la souveraineté est diffuse et dans lequel ni la censure ni l'anarchie n'ont leur place. Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission spéciale constituée sur ce texte, vous en dira plus dans quelques minutes. La France doit également être un moteur de la défense des valeurs fondamentales qui nous unissent. C'était la quatrième priorité définie par la Suède pour sa présidence du Conseil de l'Union européenne. Nous devons rester conscients de l'équilibre instable sur lequel repose la démocratie, surtout lorsqu'elle est confrontée à une importante montée des extrémismes à l'échelle de notre continent.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, à l'origine, l'Union européenne était une entente entre des nations respectueuses de leur souveraineté. Malheureusement, elle est devenue une fédération qui impose une véritable dictature idéologique, y compris pour ce qui concerne les affaires strictement intérieures des États. Il est ainsi scandaleux que, au sein de l'Union européenne, quelques pingouins veuillent empêcher la Hongrie de présider le Conseil européen, alors que c'est son tour

est pratiqué à l'encontre de la Pologne pour l'obliger à modifier son système judiciaire, lequel pourtant ne relève que de la Pologne et ne concerne que la Pologne Dans un autre domaine, la guerre en Ukraine, dans laquelle nous sommes quasiment des cobelligérants, nous coûte horriblement cher. L'explosion du prix du gaz et des matières premières, ajoutée aux aides militaires et aux subventions colossales versées à l'Ukraine, est à l'origine d'une inflation galopante et d'un endettement sans précédent. Cela pénalise lourdement les familles françaises et ruine notre pays. Je n'ai aucune hostilité contre l'Ukraine ni contre la Russie. En revanche, je tiens à dire que les vrais responsables de cette guerre sont les États-Unis, l'Otan et l'Union européenne. C'est l'impérialisme américain, conjugué à l'expansionnisme de l'Union européenne. Celle-ci n'a de cesse de s'étendre vers l'est, au détriment de la zone d'influence de la Russie. Quant à l'Otan, il aurait fallu immédiatement la dissoudre lorsque l'URSS et le pacte de Varsovie ont explosé. On veut nous faire croire que la Russie serait une menace pour la France, mais c'est un gigantesque mensonge Si la France et l'Union européenne avaient laissé la Russie tranquille, sans chercher à l'encercler, nous n'aurions eu ni cette guerre ni les difficultés économiques que nous connaissons actuellement. N'oublions pas que le coût pour la France de notre engagement dans cette guerre est égal à huit fois le montant des économies qui ont prétendument motivé la récente réforme des retraites.

Madame la

Rien, hélas, ne permet à ce stade d'entrevoir une sortie rapide du conflit. Il est en effet difficile de savoir si la contre-offensive menée par Kiev depuis un peu plus de dix jours triomphera. L'armée russe oppose pour le moment une résistance relativement solide- peut-être avait-elle été sous-estimée au regard des erreurs commises jusqu'alors par ses chefs. Dans ces conditions, on ne peut que continuer à soutenir les actions déployées par l'Union européenne depuis le début de l'agression russe. L'Europe doit en effet L'Europe doit en effet poursuivre sa mobilisation dans plusieurs directions. J'évoquerai tout d'abord le soutien aux forces armées ukrainiennes. L'Union européenne a déjà fait beaucoup, mais le passage d'une posture défensive à une stratégie offensive va mettre à rude épreuve les matériels livrés. Les stocks des armées européennes se réduisent.

Comme chacun sait, ce sont aussi les intérêts des pays européens en matière de sécurité et de défense qui sont en jeu au travers de la guerre en Ukraine. Face à cette situation, le RDSE est bien entendu favorable à la poursuite de l'aide aux forces ukrainiennes. La livraison en urgence de munitions sol-sol et de munitions d'artillerie, permise dans le cadre du fonds de la Facilité européenne pour la paix, démontre la cohésion de la très grande majorité des États membres en faveur de cette politique de soutien. Quelles sont les prochaines étapes, madame la secrétaire d'État, pour que l'approvisionnement européen en équipements militaires tienne sur le moyen et long terme ? Quoi qu'il en soit, il est certain qu'il serait difficile pour l'Europe de faire face à un autre conflit de cette intensité à ses portes. Aussi, bien que le groupe RDSE ait un temps exprimé l'idée qu'il fallait d'abord approfondir le projet européen avant de l'élargir, il apparaît aujourd'hui que le contexte géopolitique nous commande de changer de paradigme. La Communauté politique européenne, voulue par le Président de la République, est donc une bonne chose, mais elle ne suffira pas à contrer l'impérialisme russe. L'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne est bien entendu conditionnée au retour de la paix. S'agissant de son voisin moldave, en tant que présidente du groupe d'amitié France-Moldavie du Sénat, je suis sensible à son sort. Le principe consistant à maintenir des États tampons aux frontières de l'Europe me semble périmé, du fait des violations par Moscou de l'intégrité de certains de ces territoires. Aider les pays de l'Est à intégrer un ensemble démocratique doit faire partie de la boussole stratégique de l'Union européenne, au bénéfice de leur sécurité, mais aussi de la nôtre. Je vous saurais donc gré, madame la secrétaire d'État, de nous indiquer quelles perspectives d'élargissement la France envisage de défendre, et dans quelles conditions Au prochain Conseil européen, il sera également question de politique économique. Même si l'Union européenne relève la tête, les conséquences du conflit ukrainien sur les prix se font encore sentir. Lors du Conseil européen de mars dernier, il a été rappelé quelques-uns des grands axes sur lesquels l'Union européenne doit se concentrer pour renforcer sa compétitivité et sa résilience réduire ses dépendances stratégiques, en investissant dans les compétences de demain et en adaptant sa base économique, industrielle et technologique pour les transitions écologique et numérique, mais aussi approfondir le marché unique, par la suppression de certains de ses obstacles.

Avec la flambée des taux d'intérêt, la question de la dette devient de plus en plus prégnante, alors que nous devons affronter un défi de taille, celui de la décarbonation de l'économie, qui nécessite des investissements colossaux. Ne pourrait-on pas imaginer la création d'une dette environnementale, pour chacun des États membres, qui serait soustraite de l'application de critères de type Maastricht ? Enfin, on peut entendre la nécessité pour l'Europe de lever les obstacles internes au marché unique si, dans le même temps, les politiques sociales convergent davantage. Un pas vient d'être franchi avec l'accord des Vingt-Sept sur les travailleurs des plateformes, qui instaure une règle de présomption de salariat. C'est une avancée sociale qui s'ajoute à celle qui est relative aux travailleurs détachés. Il reste de nombreux domaines dans lesquels les règles d'uniformisation mériteraient d'être amplifiées. Je pense en particulier aux règles fiscales, sur lesquelles l'Union européenne manque d'élan du fait de la règle de l'unanimité. Je rappellerai qu'il a fallu en passer par un accord international pour que l'Union européenne accepte un impôt minimum commun sur les multinationales. Mes chers collègues, sur tous ces points, il s'agit en somme de rappeler que l'Europe doit tout autant renforcer sa résilience économique, pour peser à l'extérieur, qu'encourager à l'intérieur de ses frontières l'esprit de solidarité qui est au fondement du projet européen.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, tous les experts s'accordent pour dire que nous sommes entrés dans une ère multicrises covid-19, guerre en Ukraine, événements climatiques, crises économiques, la liste continuera sans nul doute de s'allonger. Face à ce constat, l'Union européenne, habituellement si prompte à se reposer sur les capacités d'autorégulation du marché, s'est décidée depuis quelques années à changer de doctrine. Elle cherche à adapter ses règles pour mieux faire face à ces bouleversements.

par la Commission européenne témoigne d'une volonté de mieux gérer en amont les risques, mais nous sommes encore loin d'avoir atteint cet objectif. Les divergences d'intérêts des Vingt-Sept et le manque de ressources propres ne nous aident pas à atteindre l'ambition de rapidité et d'efficacité que l'Union européenne affiche. C'est notamment le cas en matière de sécurité et de souveraineté économique, sujet à l'ordre du jour du prochain Conseil européen. Je ne nie pas que de belles avancées aient été obtenues en la matière, qu'il s'agisse de plan RePowerEU, du, du plan industriel du Pacte vert, de l'instrument anti-subvention ou encore de l'accélération des projets importants d'intérêt européen commun

doté d'un montant de 400 milliards de dollars, vise à faire enfin entrer le pays dans une ère écologique, mais en favorisant les entreprises américaines à grands coups de subventions publiques et de crédits d'impôt. Je ne cherche pas à être défaitiste en disant cela. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a lui-même reconnu l'insuffisance des mesures européennes. Il a ainsi déclaré : « Ce que nous avons fait n'est pas suffisant au niveau européen. Il faut avec beaucoup plus de force et avec des instruments financiers beaucoup plus puissants défendre notre industrie européenne. Face aux risques commerciaux, aux menaces de délocalisation d'entreprises du vieux continent vers les États-Unis et à la perte de notre avance technologique en matière d'écologie, l'Europe s'est réveillée, mais bien tard. Qui plus est, les Vingt-Sept se déchirent sur la méthode, en particulier quant à la possibilité d'accorder des subventions publiques

Enfin, les pays de l'Est sont inquiets de ne pas pouvoir suivre les pays qui disposeraient de plus de moyens qu'eux pour subventionner les entreprises ; ils redoutent qu'une course aux aides ne se mette en place en Europe.

aura été définitivement achevé, car l'afflux d'investissements privés ne pourra se produire efficacement que s'il existe de vastes réserves de capitaux privés attendant d'être investis, ce qui manque actuellement dans l'Union

Il serait alors possible, par exemple, de mieux contrôler les investissements réalisés dans des pays tiers, de réformer les conditions d'accès aux marchés publics en favorisant les entreprises implantées dans l'Union européenne ou encore de réviser les droits de douane pour les importations en provenance Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières constitue d'ailleurs un premier pas dans le sens d'une préférence communautaire, de même que le règlement relatif aux subventions étrangères faussant le marché intérieur. Il semblerait donc logique de continuer dans cette voie tout en allant plus loin. J'admets que l'équilibre est difficile à trouver, entre préservation des intérêts des vingt-sept États membres et nécessité de ne pas créer de conflit commercial avec des pays tiers. La préférence européenne me semble toutefois une piste intéressante à explorer dans la mesure où un fonds de souveraineté pourrait devenir un simple échelon supplémentaire des Piiec et perdre ainsi toute valeur ajoutée.

j'ajouterai qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui devrait nous guider : réagir rapidement et efficacement face à des risques économiques. N'oublions pas que le plan chinois a sept ans et que l'IRA existe depuis bientôt un an. Nous devons faire en sorte de disposer de nouveaux outils pour défendre nos industries européennes dans les meilleurs délais. À ce stade, la Commission européenne semble chercher non pas à construire une réelle stratégie, mais seulement à ouvrir une réflexion sur la thématique de la sécurité économique. Nous comptons donc sur le Gouvernement pour plaider en faveur d'une accélération du processus. La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

L'honnêteté oblige à dire que non. Aucune voie légale n'aurait permis à ces gens d'espérer pouvoir rejoindre leur famille en Europe.

de la mer et de leur engagement à accueillir les bateaux de naufragés et de sauvetage en mer. Bien entendu, cela passe par une réforme du règlement de Dublin d'une autre ampleur que ce qui est prévu

tous les abus des grandes plateformes extraeuropéennes ni certains dysfonctionnements qui sont intrinsèquement liés à leur modèle économique, à leur absence de statut, donc de vraie responsabilité.

extraeuropéennes. N'ayons pas peur des mots, il faut assumer le choix d'une préférence communautaire pour nos entreprises. Les impératifs de sécurité nationale peuvent tout à fait justifier des exemptions aux règles de l'Organisation mondiale

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de leur prochaine réunion, les chefs d'État et de gouvernement aborderont un sujet fondamental pour notre continent : l'asile et les migrations. Il semble qu'à cette occasion ils puissent enfin constater non pas seulement des divergences irréconciliables et des blocages insolubles, mais bien quelques avancées concrètes.

Il reste donc un temps finalement assez court pour clore une négociation à la fois explosive et enkystée depuis tant d'années. L'aboutissement du processus dépendra essentiellement de la capacité à régler la question qui, jusqu'à présent, a fait dérailler toutes les discussions : celle de la solidarité Malgré l'abstention de quatre pays- rien que cela ! -et l'opposition formelle de la Pologne et de la Hongrie, les États membres semblent être parvenus à s'entendre autour d'un mécanisme que l'on pourrait qualifier d'hybride et de flexible. Dans ce cadre, 30 000 demandeurs d'asile au moins devraient être relocalisés chaque année

sa mise en oeuvre soulève encore bien des questions opérationnelles, mais il a le mérite d'organiser une forme de solidarité alternative à la relocalisation obligatoire

Les eurodéputés défendent l'idée selon laquelle les engagements annuels de solidarité devraient être obligatoirement constitués, à 80 % au moins, de relocalisations, le reste pouvant prendre la forme de mesures de soutien en matériel ou en personnel.

Ajoutons à cela qu'après l'épisode lié à la fin des moteurs thermiques en Europe le caractère hétéroclite de la coalition allemande se rappelle une nouvelle fois à notre bon souvenir. Les Verts allemands, rejoignant leurs homologues européens et une partie des sociaux-démocrates, ont ainsi d'ores et déjà fait savoir sans équivoque qu'ils s'opposeraient au compromis trouvé de haute lutte par les États membres. Je note avec intérêt que les institutions européennes semblent enfin avancer sur la question fondamentale, existentielle même, de l'asile et de l'immigration.

elle ne peut en aucun cas se permettre le luxe d'une nouvelle législature pour rien sur cette question ; elle doit donc au plus vite maîtriser réellement ses frontières. Quant à la France,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, lors de leur réunion du 29 et du 30 juin prochain, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne vont devoir traiter d'un ensemble de sujets qui concernent tous trait, peu ou prou, la situation et le positionnement de l'Union européenne dans un environnement géopolitique particulièrement difficile, ainsi que sa capacité, dans ce contexte, à préserver ses intérêts et affirmer ses valeurs.

sans paraître toutefois faire la moindre concession sur le droit de l'Ukraine à recouvrer l'intégralité de son territoire national. Il faut espérer, en tout cas, que l'admirable cohésion dont ont fait preuve les États membres de l'Union jusqu'à présent ne commencera pas à se fissurer. L'approbation d'un onzième paquet de sanctions européennes contre la Russie fait, à cet égard, figure de test. Les propositions de la Commission, récemment débattues, reposent sur une préoccupation légitime : celle d'éviter que les nombreuses sanctions déjà adoptées ne soient contournées par la Russie avec la complicité de pays

à certains éléments importants du paquet, tandis que l'Allemagne fait, une fois de plus, montre de frilosité à l'égard de tout ce qui pourrait contrarier la Chine et remettre en cause les fructueuses relations commerciales qu'elle entretient avec ce pays.

européen sera par ailleurs invité à se pencher sur les futures réparations par la Russie des dommages de guerre causés à l'Ukraine et sur la mobilisation à cette fin des avoirs russes gelés en Europe. Ces questions pourraient sembler prématurées à certains, mais j'estime que, outre le souci des intérêts fondamentaux de l'Ukraine, ses alliés européens doivent aussi avoir celui de ne pas se faire exclure par d'autres du grand chantier de reconstruction qui ne manquera pas de s'ouvrir une fois le conflit terminé. Les possibilités économiques offertes devront être à la mesure des efforts consentis par notre pays dans les domaines militaire, diplomatique, financier et humanitaire. En ce qui concerne la perspective européenne de l'Ukraine,

tenir compte du fait que d'autres pays figurent déjà sur la liste d'attente et que notre opinion publique, en l'état actuel des choses, n'est pas favorable à un nouvel élargissement. l'un des effets de la guerre en Ukraine a été de relancer le débat sur la politique commune de sécurité et de défense et sur la coopération entre l'Union européenne et l'Otan. En cohérence avec la boussole stratégique, adoptée l'année dernière par le Conseil

il convient d'éviter que les efforts budgétaires notablement accrus de plusieurs États membres en matière de défense ne profitent aux fournisseurs des pays tiers. une discussion sur les questions de migrations est prévue à l'agenda du Conseil européen. Elle est évidemment indispensable pour progresser enfin sur cette question très sensible. Faute de s'entendre sur des quotas ou des mécanismes de répartition des migrants, nos pays doivent au moins unir leurs efforts pour organiser le renvoi effectif des migrants clandestins et des déboutés du droit d'asile vers leur pays d'origine. Cela implique de mettre la pression sur les pays concernés, notamment ceux de la rive sud de la Méditerranée, par tous les moyens à la disposition de l'Union européenne : octroi de visas, préférences commerciales, aides financières

Il est attristant, à la lecture de ces documents, de constater que la France est, encore une fois, pointée du doigt pour des déséquilibres macroéconomiques importants, une dette publique excessive et insoutenable « à moyen terme », des problèmes sérieux de compétitivité et une faible progression de la productivité du travail. Par ailleurs, les réformes structurelles nécessaires pour remettre en ordre les finances publiques à plus long terme sont considérées comme insuffisantes à ce stade, et des doutes sont émis sur la capacité du Gouvernement d'en entreprendre de nouvelles. Ce diagnostic et les recommandations dont il est assorti sont évidemment à prendre très au sérieux, non pas parce qu'ils émanent des institutions européennes, mais parce qu'il y va de l'intérêt et de la crédibilité de notre pays et de sa capacité à faire face à tous les défis qui se présentent à lui.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 29 et le 30 juin prochain, le Conseil européen se réunira. Il y sera question de la politique économique de l'Union européenne, au travers des conclusions du Conseil sur la politique industrielle et sur le marché unique, ainsi que sur la compétitivité et la productivité à long terme de l'Europe. La situation économique, la sécurité et la résilience économique de l'Union C'est sur ces points que je souhaite m'attarder, car il me paraît nécessaire de faire entendre la voix de la France. Par son histoire, sa longue tradition industrielle et sa vision gaulliste d'une économie au service de la souveraineté nationale, la France a des valeurs dont l'Union européenne doit pouvoir s'inspirer. Depuis trop longtemps, nos gouvernants européens me semblent faire montre d'une certaine naïveté dans leur vision des rapports de force économiques mondiaux. Nous en portons collectivement la responsabilité, quelle que soit notre tendance politique ou notre nationalité. Au tournant des années Maastricht, notre croyance dans un marché mondial porteur de toutes les vertus était solidement ancrée. Confiants dans notre potentiel économique, nous croyions que les échanges mondiaux ne pourraient pas nous être Dans une sorte de surinterprétation de la théorie des avantages comparatifs, l'économie européenne s'est transformée, passant d'une économie industrielle à une économie de service. Le marché étant le remède à tout et ne pouvant nous nuire, pourquoi garder ces grandes usines laides et polluantes quand on pouvait faire fabriquer ailleurs ? Le concept même de souveraineté semblait appartenir à un autre temps. Cette vision essentialisée du marché nous a considérablement affaiblis, alors que se réveillaient des géants économiques et que d'autres, outre-Atlantique, renforçaient leurs armes dans la concurrence mondiale. Depuis, la crise sanitaire et la crise ukrainienne ont remis au goût du jour le concept de souveraineté économique, voire la question d'une souveraineté européenne. Le chemin à parcourir est encore long.

À l'inverse de l'Union européenne, ces puissances concurrentes contrôlent la chaîne de production de bout en bout. De l'extraction des terres rares à la production des batteries, puis à l'assemblage des véhicules, nos constructeurs font face à une concurrence puissante et inquiétante. il s'agit non pas d'avantages technologiques, mais bien de la capacité d'industries étrangères à mobiliser des moyens et des ressources immenses pour conquérir de nouveaux marchés. préoccupant que ces industries concurrentes proviennent parfois de pays ne pratiquant malheureusement ni embargo ni sanctions à l'égard de la Russie. Elles continueront donc d'avoir accès aux ressources minières russes, nos industriels européens devront se fournir ailleurs à prix d'or et n'auront pas d'autre choix que de reporter le coût supplémentaire sur les consommateurs. D'une politique économique naïve et mal préparée découlent des conséquences sociales qui distendent le lien démocratique entre l'Europe et ses citoyens. Les zones à faibles émissions (ZFE) en sont un bon exemple

D'une Europe pourvoyeuse d'un marché unique laissant librement circuler les individus et les biens, sans frontières ni barrières douanières, nous risquons de nous retrouver dans une situation ou l'octroi à l'entrée des villes dernier point concerne la question énergétique. Entre atermoiements, ordres et contre-ordres, la politique de l'Union européenne mérite d'être débattue. Le temps imparti est malheureusement trop court pour revenir sur le projet Hercule prévu pour EDF, sur le mécanisme européen de couplage des prix de l'électricité sur celui du gaz ou encore sur le label vert

Une fois encore, nous fixons des objectifs qui ne sont atteignables qu'avec le concours d'industries étrangères, et souvent au prix d'une déstabilisation de notre propre filière. En effet, nous importons actuellement entre 70 % et 80 % des équipements nécessaires à la production d'énergies renouvelables. Les filières scandinaves et allemandes peinent à rivaliser avec leurs concurrents asiatiques. face à des entreprises qui disposent à domicile des ressources nécessaires à la fabrication des équipements : terres rares, métaux critiques, etc. Sans compter qu'il s'agit là de futurs déchets pour le traitement desquels les filières de recyclage européennes sont balbutiantes et déjà convoitées par la concurrence internationale. Madame la secrétaire d'État, mes collègues vous ont déjà posé de nombreuses questions. Aussi, pour conclure, je dirai simplement que l'Union européenne continue parfois de prendre pour elle-même des décisions économiques qui font le jeu d'intérêts étrangers et qui éloignent démocratiquement le citoyen européen. Elle doit veiller à faire émerger une souveraineté européenne sans empiéter sur celle des États membres, et bâtir une politique économique et environnementale forte.

nous veillerons évidemment, lors de l'examen du texte, à préserver à la fois nos intérêts de sécurité nationale et la répartition des compétences qui est prévue par les traités.

J'ai également été interrogée sur l'adoption du onzième paquet de sanctions, qui est prévue pour le prochain conseil des ministres des affaires étrangères de l'Union européenne le 26 juin prochain. Il comporte deux volets le premier, sur la mise en oeuvre d'un mécanisme anti-contournement des sanctions, pour s'assurer de l'efficacité de celles-ci, le second, sur l'ajout d'une centaine de désignations individuelles contre des responsables russes

de la France. Venons-en à l'économie. Monsieur le sénateur Raynal, vous m'avez interrogé sur la révision du cadre financier pluriannuel et la réforme de la gouvernance économique européenne, dont le contenu, comme vous le savez, a été communiqué par la Commission européenne aujourd'hui même.

l'instauration d'un contrôle des prises de participation et des investissements dans les secteurs stratégiques. Sur la gouvernance économique,

numérique. Nous regrettons que la proposition d'avril réintroduise des règles numériques automatiques, car elles se sont révélées procycliques dans les années précédentes. Il nous semble important de préserver l'esprit des réformes, ce qui inclut bien sûr la soutenabilité des finances publiques. Ces règles numériques

cette optique que la France entretient un dialogue nourri avec Tunis. Le Président de la République va ainsi s'entretenir avec le président Saïed en marge du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. De plus, nous nous mobilisions auprès de nos partenaires européens pour soutenir la Tunisie Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni et Mark Rutte s'y sont ainsi rendus le 12 juin dernier pour annoncer un paquet global de soutien que nous avons contribué à élaborer et dont nous approuvons les orientations.

Elle a été rappelée la semaine dernière par le ministre délégué chargé du commerce extérieur, Olivier Becht : nous ne pouvons pas accepter l'accord en l'état. Comme je le dis à tous nos partenaires européens, cet accord doit être complété par des engagements additionnels contraignants et ambitieux sur le développement durable. L'accord de Paris doit en être une clause essentielle, et l'accord avec le Mercosur doit être aligné avec la nouvelle approche de l'Union européenne en matière de commerce et de développement durable. Nous portons cette position auprès de la Commission

le plus vite possible. C'est indispensable pour protéger les consommateurs, pour lutter contre la volatilité des prix et pour encourager les investissements dans les énergies décarbonées. Nous travaillons en ce sens.

au travers d'un cadre de régulation qui promouvra le modèle et les valeurs européens dans le domaine du numérique, auprès de nos partenaires et de manière multilatérale, avec le même succès, je l'espère, que pour le